Conformément aux dispositions de l'article L. 567-1 du code électoral, la commission des lois a fait connaître qu'elle a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 28 voix pour, 3 voix contre -à la nomination par le président du Sénat de M. Michel Sappin aux fonctions de membre de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. L'ordre du jour appelle la discussion, à la demande du relative à l'aménagement du permis à points dans la perspective de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure sur le réseau secondaire, présentée par Mme Sylvie Goy-Chavent et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, auteur de la proposition de loi.

la proposition de loi relative à l'aménagement du permis à points entame son parcours parlementaire dans le cadre de la niche réservée au groupe Union Centriste, sans lequel ce texte n'aurait jamais été soumis au vote.

et le permis à points, alors que près de cent dix sénateurs ont cosigné cette proposition de loi. Je le regrette. Comme vous le savez, depuis son annonce, le 9 janvier 2018, dans le cadre d'un grand plan de sécurité routière, l'abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 80 kilomètres par heure cristallise l'opposition d'une majorité des automobilistes et de très nombreux élus locaux. Rappelons que la décision du Gouvernement a été prise sans aucune concertation ni avec les associations d'automobilistes, ni avec les conseils départementaux- pourtant gestionnaires des routes -, ni avec les parlementaires. Malgré de très vives protestations, cette Malgré de très vives protestations, cette mesure a donc été imposée aux Français le dimanche 1 juillet dernier. Il n'est pourtant pas du tout certain qu'Emmanuel Macron ait été élu à la présidence de la République pour cela. Peut-être en paye-t-il un peu le prix Maire d'une commune rurale pendant plus de vingt ans, au contact direct de mes concitoyens, j'ai très vite compris que le Gouvernement commettait une grave erreur en imposant les 80 kilomètres par heure et j'ai tenté d'alerter le Président de la République, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur.

sincèrement. Cette proposition de loi a le mérite d'ouvrir le débat essentiel de l'équilibre à trouver en matière de sécurité routière. Le permis à points s'inscrit dans un cadre préventif et pédagogique, son but est d'inciter les usagers de la route à modifier leur comportement. Je suis la première à reconnaître que, malgré d'incontestables progrès, la mortalité routière demeure un fléau dans notre pays. Chaque année, des milliers de vies sont brisées et des milliers de familles sont détruites. À travers cette proposition de loi, il ne s'agit en aucun cas pour moi de remettre en cause la légitimité du permis à points et encore moins d'encourager des comportements à risque sur nos routes. Le Gouvernement nous assure que l'abaissement de la vitesse à 80 kilomètres par heure a fait baisser la mortalité routière. C'est faux ! Je souhaite de tout coeur que ce soit effectivement le cas.

Les cadres de La République En Marche sont intelligents- de leur propre aveu, ils le sont même trop pour nous -, mais, en vérité, ils n'ont souvent aucune expérience politique, aucune expérience de terrain et sont complètement déconnectés de la vraie vie des Français. Mes chers collègues, on ne fait pas de la politique avec des chiffres, on fait de la politique avec le coeur quand on aime les Français, quand on aime la France. J'invite donc le Gouvernement à penser aux dizaines de millions de Français qui habitent les zones rurales ou périurbaines et qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture chaque jour pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour emmener leurs enfants à l'école, à la crèche, etc. Dans ces zones, il n'y a pas d'alternative.

pour aller travailler, qui a le goût de l'effort, cette France des campagnes et des périphéries urbaines, cette France trop souvent méprisée et qui se sent aujourd'hui abandonnée.

C'est de cela que nous parlons aujourd'hui et pas d'autre chose. Sommes-nous sourds aux appels des Français ? Ne sont-ils pas assez nombreux à défier nos institutions sur les ronds-points et à détruire les radars sur le bord des routes ? Que devront-ils faire encore pour que nous les écoutions enfin ? N'en déplaise au Gouvernement, les automobilistes français ne sont pas tous des délinquants, ce sont des citoyens intelligents qui ont compris l'effet pédagogique du permis à points, mais qui en ont assez de se sentir piégés, voire humiliés, et, en tout état de cause, pas entendus ou mal représentés. Tous n'ont pas les moyens de s'offrir des stages de récupération de points ou des chauffeurs. Ce qui est en cause, ce n'est pas la politique de sécurité routière, c'est le sentiment d'injustice qui gangrène notre pays. Comment voulez-vous être ferme si vous n'êtes pas juste, monsieur le secrétaire À force de toujours taper sur les automobilistes, le Gouvernement est-il juste ? Avant de faire passer des mesures répressives au forceps, j'aurais souhaité que le Gouvernement annonce un plan massif d'investissements sur le réseau secondaire,

Je profite de cette prise de parole pour évoquer ici les centaines de milliers de faux permis étrangers qui circulent dans notre pays. On dit que 5 % à 10 % des permis de conduire sont des quand les conducteurs ont un permis ! -, mais aucun ministre ne monte à la tribune de cet hémicycle ou ne se rend au 20 heures pour parler de cela ! Une collègue sénatrice me disait hier que ma proposition de loi ne servait à rien. Ma foi, nous verrons ; les Français jugeront. Comment voulez-vous que la colère ne monte pas dans notre pays ? En rédigeant ce plaidoyer, j'ai fait quelques recherches et j'ai constaté que le permis à points avait été instauré par la loi du 10 juillet 1989.

Je voudrais seulement démontrer la nécessité de répondre à la colère qui monte dans le pays et qui deviendra très vite incontrôlable. Aménager le permis à points ne la fera pas taire, je vous l'accorde, mais voter en faveur de ce texte serait un très bon signal adressé à nos concitoyens et le Sénat en sortirait grandi. Pour les dépassements de vitesse entraînant la perte d'un seul point, pourquoi ne pas permettre à nos concitoyens de récupérer ce point à l'issue d'une période de trois mois au lieu de six mois actuellement, sous réserve, bien sûr, qu'ils n'aient commis aucune nouvelle infraction

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur une proposition de loi, déposée par Mme Sylvie Goy-Chavent et plusieurs de nos collègues, relative à l'aménagement du permis à points dans la perspective de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure sur le réseau secondaire. Ce texte s'inscrit dans un contexte que nous connaissons tous et dont nous avons déjà eu à débattre au Sénat : la forte incompréhension de la population à propos de l'abaissement de 90 à 80 kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. Je mesure, mes chers collègues, l'engagement de chacun d'entre vous sur cette question particulièrement sensible dans le contexte social actuel et qui nous vaut régulièrement des sollicitations de nos concitoyens. À titre de compensation de ce durcissement de la réglementation routière, les auteurs de la proposition de loi entendent alléger les sanctions appliquées aux infractions les moins graves, en assouplissant les règles de récupération de points. Le dispositif proposé, que nous a rappelé notre collègue Sylvie Goy-Chavent, est relativement simple : il consiste à réduire de six mois à trois mois le délai dans lequel les personnes ayant perdu un seul point à leur permis de conduire peuvent le récupérer, si elles n'ont pas commis, dans ce délai, de nouvelles infractions. Il s'agit, dans l'esprit des auteurs de la proposition de loi, d'éviter que le passage à 80 kilomètres par heure ne pénalise de manière démesurée les usagers de la route, en leur faisant risquer de perdre plus de points sur leur permis de conduire. Notons que quatre infractions seulement sont aujourd'hui concernées par le retrait d'un seul point : les petits excès de vitesse, inférieurs à 20 kilomètres par heure ; l'absence de port de gants homologués par les motocyclistes ; le chevauchement d'une ligne continue et le chevauchement des lignes délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sur autoroute. Pour autant, si peu d'infractions sont concernées, le champ d'application de la proposition de loi serait assez large, car plus de la moitié des points qui sont chaque année retirés le sont pour de petites infractions au code de la route. En 2017, par exemple, sur les quelque 15 millions de points de permis de conduire qui ont été retirés, près de 9 millions l'ont été pour des infractions légères, punies du retrait d'un seul point.

Une mesure qui n'est pas acceptée ne sera que peu respectée, c'est d'ailleurs la position que nous avions défendue, avec Michel Raison et Michèle Vullien, dans notre rapport d'information sur le passage aux 80 kilomètres Dans ce contexte, il paraît donc essentiel de s'interroger, comme le font les auteurs de la proposition de loi, sur la manière de lutter efficacement contre la délinquance routière, sans pour autant que les mesures adoptées soient jugées injustes et pénalisantes pour les usagers de la route les plus vertueux. Cette même interrogation a d'ailleurs conduit le Gouvernement à lancer récemment une réflexion sur la valorisation des comportements responsables sur la route. Une étude sur le sujet a été confiée au Conseil national de la sécurité routière son président, Yves Goasdoué, que nous avons reçu en audition, nous a indiqué que les conclusions de ce rapport seraient prochainement remises. Plusieurs propositions sont envisagées, parmi lesquelles l'idée d'introduire une forme de sursis sur le retrait de points.

La première est que la réduction de la durée de récupération de points pourrait constituer un signal négatif en matière de lutte contre l'insécurité routière. Il existe en effet un risque important que les conducteurs, certains de récupérer leurs points plus rapidement, adoptent des comportements à risque. La durée de six mois est déjà courte, si nous la réduisons, nous risquons de nuire à la vertu pédagogique du permis à points et à son efficacité en matière de lutte contre les infractions routières. Notons d'ailleurs que les personnes qui commettent une petite infraction ne sont actuellement informées du retrait de points qu'au bout de deux mois, en raison des délais de recours et des délais techniques liés à la gestion des flux. Si nous abaissions le délai de récupération de points à trois mois, les personnes concernées se verraient informées de leur retrait d'un point et de sa récupération de manière quasiment simultanée, ce qui diminuerait assurément l'utilité de la sanction. Enfin, il est important de rappeler que la proposition de loi ne porterait pas uniquement sur les excès de vitesse commis sur les routes limitées à 80 kilomètres

La seconde raison a trait à l'utilité de la proposition de loi. Les statistiques nous montrent que les délais actuellement prévus pour la récupération de points ne sont pas disproportionnés.

La plupart des personnes concernées perdent donc leur permis en raison d'infractions lourdes au code de la route, et non de petits excès de vitesse. Dans ces conditions, réduire à trois mois la durée de récupération de points n'aurait que très peu d'impact sur les invalidations de permis de conduire.

qu'elle n'apportait pas de solution viable. La sécurité routière, nous le savons tous, est une matière complexe et ses enjeux sont trop importants pour adopter des dispositions à la légère je rappelle que plus de 3 500 personnes perdent encore la vie chaque année sur la route. Il paraît dès lors préférable de conditionner toute évolution législative du permis à points à la conduite d'une étude d'impact approfondie, afin de garantir l'efficacité des mesures proposées et d'éviter tout effet de bord. Je ne doute pas, d'ailleurs, que la réflexion actuellement menée par le Conseil national pour la sécurité routière contribuera utilement à ce débat.

a fait preuve, la semaine dernière, à l'occasion du lancement du grand débat national, d'une certaine ouverture à l'égard de la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure. Il n'a pas exclu, au vu de l'incompréhension d'une grande partie de la population, de revenir sur cette mesure mise en place de manière généralisée et sans aucune concertation locale. Plutôt que d'adopter des dispositions de compensation, restons donc fidèles à la position du Sénat et continuons à soutenir l'ouverture de concertations au niveau des départements en vue d'adapter la réduction des vitesses aux réalités de chaque territoire. Pour l'ensemble de ces raisons et tout en reconnaissant l'intérêt du débat soulevé, je vous invite, au nom de la commission des lois, à ne pas adopter cette proposition de loi.

de loi dont nous débattons aujourd'hui vise à aménager le système de retrait de points sur le permis de conduire en fonction de la gravité des infractions commises par le conducteur. Avant d'évoquer devant vous le contenu de ce texte, je souhaite apporter des éléments de contexte et rappeler que le mouvement continu de baisse de la mortalité routière, constaté depuis 2003, a marqué le pas entre 2014 et 2017. Le nombre de morts liés à l'accidentalité routière est resté stable au cours de ces dernières années, à un niveau trop élevé, trop élevé, insupportable pour l'ensemble de la société française. Or, nous le savons, l'essentiel de la mortalité enregistrée intervient sur le réseau routier secondaire. Afin de faire reculer ce phénomène, le Gouvernement a pris un ensemble de décisions au cours du comité interministériel de la sécurité routière réuni en janvier 2018.

L'analyse du bilan de cette mesure devrait être communiquée par le Gouvernement de façon imminente. Je puis vous indiquer, ainsi que je l'ai fait hier à l'occasion des questions d'actualité au Gouvernement, que la tendance est positive, si l'on se borne à constater, en première analyse, les baisses de la mortalité enregistrées depuis le 1 juillet, par rapport aux mêmes mois en 2017. Il convient d'ailleurs, à ce titre, de souligner que l'augmentation massive des dégradations

Pour en revenir à l'objet de cette proposition de loi, je souhaite rappeler que les conducteurs qui commettent un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure sur les routes où la vitesse maximale autorisée a été ramenée à 80 kilomètres par heure se voient sanctionnés par le paiement d'une amende et le retrait d'un point. Cette sanction respecte le principe de proportionnalité appliqué en matière de permis à points. En effet, le nombre de points retirés sur le permis de conduire varie en fonction du niveau de dépassement de la vitesse : il est de deux points pour un dépassement compris entre 20 et 30 kilomètres

Dans ce dernier cas, l'infraction est constitutive d'une contravention de cinquième classe et sa récidive matérialise le délit de grand excès de vitesse. L'exposé des motifs de cette proposition de loi met en avant la différence que ferait naître l'abaissement à 80 kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, dans le traitement des infractions, selon que celles-ci aient été commises en zone rurale

puni d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, d'un même dépassement de vitesse en agglomération, sanctionné, quant à lui, d'une amende de quatrième classe. Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de restitution du point perdu à la suite d'une infraction pour laquelle ce retrait est

En 2017, plus de 6 millions de restitutions d'un point au terme d'une période de six mois ont été effectuées, contre seulement 5,3 millions en 2016. Le nombre de restitutions d'un point a donc augmenté de près de plus de 13 % entre ces deux années. Réduire encore ce délai serait incohérent, à nos yeux, avec les objectifs de la sécurité routière. À cet égard, il convient de nouveau de rappeler que c'est dans les zones rurales que la mortalité est la plus élevée. En outre, les retraits successifs d'un point non restitué demeurent une cause marginale d'invalidation du permis de conduire. Ainsi, malgré la règle de cumul des contraventions prévue par l'article 132-7 du code pénal, seulement 121 personnes en France ont vu leur permis de conduire invalidé en 2017 pour solde nul en n'ayant commis qu'un seul type d'infraction : des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres

revanche, cela pourrait avoir des effets psychologiques importants, dont nous ne pouvons présumer, mais qui risquent d'amener certaines personnes à faire moins attention à leur vitesse sur la route. Enfin, la gestion du permis à points, mise en oeuvre par le système national des permis de conduire, est soumise au délai d'enregistrement des infractions, qui est en moyenne de deux mois. En réduisant le délai de restitution du point à trois mois, l'usager pourrait avoir connaissance du retrait d'un point et de sa restitution pratiquement simultanément. Ce dispositif retirerait par conséquent tout l'intérêt pédagogique souhaité par le législateur dès 1992, qui est rappelé, à juste titre, dans l'exposé des motifs de la présente proposition de loi. Pour conclure, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, croyez bien que l'objectif du Gouvernement n'est pas de mettre des bâtons dans les roues aux Français,

Elle fera l'objet d'une évaluation et sera discutée au cours du grand débat, car la mobilité se situe au coeur des préoccupations de nos concitoyens, en particulier de ceux qui résident en zone rurale et qui, au quotidien, empruntent les 400 000 kilomètres

induits, sur les temps de déplacement, la cohabitation entre les poids lourds et les véhicules particuliers, la consommation de carburant ainsi que la production de CO2.

À cet égard, l'avis des présidents de conseil départemental sera essentiel. Le cas échéant, ainsi que le Président de la République l'a rappelé, le dispositif pourra être aménagé.

sur leurs tablettes au fichier des permis de conduire afin de vérifier l'usage éventuel de faux documents. Une expérimentation est en cours pour étendre cette utilisation aux polices municipales.

par heure est fléchée vers des investissements importants en milieu hospitalier, justement pour accueillir les grands blessés de la route. Enfin, je terminerai en disant que nous entendons la colère de la population, nous entendons la colère de la population, de la même façon que nous entendons aussi la colère sourde des familles de victimes auxquelles nous devons aller annoncer le décès de l'un des leurs sur la route à cause de vitesses excessives. C'est aussi une colère qu'il faut savoir entendre ! Encore une fois, le grand débat permettra

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en signant les lettres patentes royales de 1552 ordonnant de planter des ormes le long des voiries, Henri II ne se doutait pas que, quelques siècles plus tard, cette décision pourrait être remise en cause pour des questions de sécurité. Il était à l'époque question de préserver les chemins contre le grignotage par les cultures et, plus tard, d'offrir une ombre confortable aux usagers estivaux des routes ou de retenir la poussière soulevée par les véhicules sur les routes qu'on appelait à l'époque « blanches Les premières réglementations concernant le réseau routier se sont donc inscrites dans une pure logique d'aménagement du territoire. L'objectif était alors de répondre aux « besoins de chacun ». Cette ambition routière a eu sa part dans le processus historique d'unification de notre pays. de notre pays. La préoccupation de sécurité routière est relativement récente. Nous avons d'abord cherché à gagner en vitesse. Pour cela, nos voitures se sont mécanisées, sont devenues plus puissantes, ce qui était alors une fierté nationale. Faut-il rappeler que le premier congrès international de l'automobile de 1900 s'est tenu à Paris ? En parallèle de ces évolutions technologiques, les Français sont devenus « averses au risque Le développement concomitant du secteur de l'assurance en témoigne. Tant et si bien que ce sont plus les motifs de sécurité routière qui menacent aujourd'hui les arbres le long de nos routes que l'invention du goudronnage, de la climatisation, ou le chancre doré. C'est le même objectif de sécurité routière qui a présidé à la parution du décret du 15 juin 2018 prévoyant l'abaissement de la vitesse maximale de 90 à 80 kilomètres par heure Depuis l'annonce de cette décision, de nombreux parlementaires ont réfléchi aux moyens de relayer les doléances des citoyens de la « France périphérique », fortement dépendants de leurs voitures. À l'Assemblée nationale, l'examen d'une proposition de loi de notre collègue député Vincent Descoeur, du Cantal, a cependant coupé l'herbe sous le pied à toute initiative parlementaire. Mme la ministre Jacqueline Gourault avait alors considéré que « la fixation des vitesses maximales autorisées sur les routes est clairement une compétence réglementaire du Premier ministre ». Fermez le ban ! C'est aussi le cas du pouvoir de modulation des autorités locales, également fixé dans la partie réglementaire du code de la route.

Dans cette attente, la volonté de relayer cette préoccupation de nombre de nos concitoyens a poussé plusieurs membres du groupe du RDSE à cosigner la proposition de loi aujourd'hui présentée par nos collègues centristes. De notre côté, nous pensons qu'un principe général devrait encadrer la fixation des vitesses maximales pour permettre une meilleure articulation des objectifs de sécurité routière et d'aménagement du territoire. Nous proposerons cette solution dans notre prochain espace réservé. soit affaiblie, il faut souligner que la sécurité routière pourrait être plus intelligemment mise en oeuvre, en associant mieux les acteurs locaux et en développant des équipements innovants. On sait qu'une grande partie des accidents sont causés par des chaussées défaillantes et qu'ils augmentent considérablement les jours de pluie. Voilà des sujets qui devraient être examinés en priorité pour réussir à passer sous la barre des 2 000 morts par an ! Nous avons entendu les critiques adressées à la disposition précise du texte de Mme Goy-Chavent. La position au sein du groupe n'est d'ailleurs pas unanime. Mais, vous le savez tous, le contournement du domaine réglementaire est souvent un exercice baroque ... Certains y verront peut-être de l'« parlementaire ». Nous qui aimons l'histoire, nous préférons y voir la conséquence directe du parlementarisme rationalisé. Cependant, la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement n'est pas des plus évidentes, surtout lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts les les plus primaires. Cette frontière est même parfois incompréhensible, y compris pour des hommes de loi. Comment expliquer que l'on trouve aujourd'hui dans la partie législative du code de la route des dispositions précises relatives à l'équipement en pneus adaptés en zone de montagne, au poids des véhicules ou à l'émission de substances polluantes, mais rien sur les limites de vitesse ? Dans ce contexte, la position majoritaire au sein du groupe est donc la suivante : si le Gouvernement propose des évolutions par décret, comme il s'y est engagé, nous le soutiendrons si le Parlement propose une disposition destinée à le pousser à prendre ces modifications, nous la voterons ! Réduire la durée de récupération d'un point de permis perdu à la suite d'un dépassement de vitesse n'est pas la solution parfaite, mais notre choix se réduit aujourd'hui à deux propositions bancales : soit l'abaissement de la vitesse sur toutes les routes de France, quelle que soit leur dangerosité soit l'atténuation de la sanction lorsque l'on déroge à cet abaissement. Faute de mieux, la majorité du groupe du RDSE choisira la seconde solution, tandis que le vote de cinq de mes autres collègues sera avant tout guidé par le souci de la clarté juridique. Ils sont en quelque sorte, madame l'auteur de la proposition de loi, sentimentalement pour le texte, mais juridiquement contre. La parole est

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus sur les critères restrictifs de recevabilité

la société d'autoroutes SANEF vient d'instaurer, à la barrière de Boulay-Moselle, un système entièrement nouveau de péage, en indiquant qu'elle avait l'intention de le généraliser partout. Or ce nouveau système est tout à fait scandaleux.

s'arrêter. Sous couvert de laisser passer les gens sans s'arrêter, la SANEF instaure un système qui supprime la possibilité pour les autres usagers de l'autoroute de payer au guichet, comme c'est le cas normalement. Ceux qui ne seront pas abonnés à ce nouveau système seront donc obligés

et je déplore que le Gouvernement cautionne une telle dérive de la part des sociétés d'autoroutes. C'est véritablement une honte et l'on se moque du monde : prétendre faciliter la vie de l'usager en faciliter la vie de l'usager en lui interdisant de payer au guichet, que ce soit par carte ou en espèces, et en l'obligeant à sortir de sa voiture, vous vous rendez compte, c'est à en écoeurer les gens ! Petit à petit, la SANEF espère que tout le monde prendra un abonnement au péage.

je tiens avant toute chose à saluer l'initiative de Sylvie Goy-Chavent. Si notre groupe a souhaité que sa proposition de loi soit inscrite aujourd'hui dans notre espace réservé, c'est parce que la problématique qu'elle aborde qu'elle aborde nous apparaît très importante, qu'elle concerne un grand nombre de nos concitoyens et qu'elle est profondément d'actualité. Plus largement, cela permet à la Haute Assemblée de débattre d'un sujet qu'elle connaît bien. En effet, les évolutions du code de la route, puisque c'est d'abord de cela qu'il est question cet après-midi, ont toujours fait l'objet d'une attention particulière du Sénat. Sur ces sujets, il a déjà été régulièrement force de proposition. Les règles du code de la route retiennent particulièrement notre attention pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est question de sécurité routière et que le nombre de morts sur nos routes reste trop important, même s'il faut se rappeler que, en l'an 2000, nous avions encore près de 8 000 morts par an sur nos routes. La deuxième raison justifiant un intérêt tout particulier pour cette matière, c'est parce qu'elle concerne quotidiennement une très large partie de nos concitoyens, qu'ils soient automobilistes, motards, cyclistes ou piétons. Ces règles intéressent tous les Français. Nous savons bien que, dès qu'il est question de les modifier, évidemment, le débat s'enflamme. Une fois n'est pas coutume, la décision du Gouvernement d'abaisser la vitesse à 80 kilomètres par heure sur les routes secondaires a suscité de vives réactions sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les territoires ruraux, les plus pénalisés. En effet, pour beaucoup, et particulièrement pour les habitants de ces territoires, la route est une habitude quotidienne. Certains passent plus d'une heure au volant pour se rendre sur leur lieu de travail le matin- pareillement le soir -, et ce sur les mêmes routes, depuis des années, à la même vitesse : 90 kilomètres par heure. Or, depuis le 1 juillet dernier, cette limitation de vitesse est réduite sur l'ensemble du réseau secondaire. On comprend ainsi aisément que de nombreux conducteurs ont pu et pourront perdre un point à cette occasion.

Le système du permis à points, en vigueur depuis 1992, indexe la gravité des infractions commises sur la sanction en vue d'inciter les conducteurs à réfléchir sur les conséquences de leur comportement sur la route. Les ruraux sont particulièrement dépendants de leur permis, et la majorité ne peut faire sans. Nous savons tous, mes chers collègues, que, dans de nombreux territoires, il n'existe aucune alternative à la voiture.

je ne prends ni le métro, ni le bus, ni le tram ! Il n'existe donc aucune alternative à la voiture. C'est d'ailleurs l'une des problématiques fondamentales qui est abordée dans le cadre du grand débat national lancé par le Président de la République. Pour les habitants de ces territoires, plus que pour d'autres, c'est un facteur de stress particulier, quand on sait qu'un petit écart de vitesse peut faire perdre un point pendant six mois. L'assouplissement que nous proposons à travers ce texte ne vise absolument pas à remettre en cause notre politique de sécurité routière ou le système du permis à points. Il n'est pas proposé d'exempter de sanctions le conducteur qui a commis une infraction grave. Il est simplement proposé de minorer les conséquences sur son permis de conduire, non pas de l'exonérer du règlement de l'amende due en cas de dépassement de la vitesse maximum autorisée. Pour reprendre les termes de l'exposé des motifs du texte, il s'agit de « limiter les effets d'une décision gouvernementale aussi inefficace qu'injuste », et en aucun cas de tendre vers une impunité du chauffard. Il s'agit aussi de montrer que le Sénat que le Sénat est à l'écoute des Français, à l'écoute des territoires et entend proposer des solutions pragmatiques. Absolument ! Je rappelle d'ailleurs que notre assemblée tente de faire entendre sa voix sur l'abaissement de 90 à 80 kilomètres par heure depuis la publication du rapport d'information de nos collègues Michel Raison, Michèle Vullien et Jean-Luc Fichet, en avril dernier ! Nous espérons que la voix du Sénat

Le Premier ministre, enfin, l'a lui-même admis : cette mesure n'est le résultat d'aucune expérimentation fiable. Plusieurs ministres s'y sont opposés, et le Président de la République aurait lui-même dit que c'était une « connerie ». Il s'agissait d'envoyer un signal fort pour que baisse de manière significative le nombre de morts. La baisse a-t-elle été significative ? Assurément non, mais l'incompréhension et le mécontentement, oui ! On le voit avec les « gilets jaunes À aucun moment le Gouvernement n'a évoqué la qualité des infrastructures routières, qui joue pourtant un rôle fondamental pour la sécurité routière. le Sénat avait pourtant donné l'alerte à ce sujet en soulignant la tendance à la dégradation du réseau routier national observée depuis quelques années.

On parle des hôpitaux : je n'y crois pas. En fait, on rembourse la dette. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi vise à faciliter la récupération de points afin de compenser le durcissement de la réglementation routière. Il est ainsi proposé que, pour les infractions ayant entraîné le retrait d'un seul point, le délai au terme duquel ce point est réattribué, si aucune infraction donnant lieu à un nouveau retrait de point n'a été commise, soit ramené à trois mois au lieu de six mois. C'est pure logique En 2011, j'ai été l'auteur de l'amendement permettant notamment la récupération d'un point en six mois au lieu d'un an. Que n'ai-je entendu de la part de M. Hortefeux, alors ministre ? C'était la révolution ! À l'époque, cette modification n'a eu aucune conséquence sur le nombre de morts. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous n'avons plus de radars en état de marche dans les territoires, détruits ou bâchés. Y a-t-il eu plus de morts ? Il ne semble pas. La généralisation des 80 kilomètres par heure aura nécessairement des conséquences sur le nombre de personnes roulant sans permis. Entre 2012 et 2017, ce chiffre a déjà augmenté de 30 % pour atteindre 600 000. Il ne faut pas oublier que, dans les territoires ruraux, il n'existe aucune alternative à la voiture. Nous ne sommes pas à Paris : il n'y a ni métro ni bus, et chacun doit se débrouiller. Les pistes évoquées dans le projet de loi d'orientation des mobilités ne seront pas opérationnelles demain. Après des mois d'obstination, si le Président de la République se dit prêt à rouvrir le débat sur des aménagements à la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure, nous n'en connaissons ni l'issue ni le délai. Pendant ce temps, l'argent rentre ! Le Sénat, lui, milite depuis un an

Dans cette attente, je suis personnellement favorable à cette proposition de loi, qui a le mérite de relancer le débat sur la politique de sécurité routière. Il appartiendra à l'État, monsieur le secrétaire d'État, de s'organiser pour que l'information du retrait de point et sa récupération ne soient pas concomitantes. Il s'agit aujourd'hui non plus d'aménager les 80 kilomètres par heure, mais de rétablir la confiance des citoyens dans la politique de sécurité routière, promouvoir des comportements raisonnables et responsables sur la route pour toujours plus de sécurité, d'instaurer le bonus de points, de distinguer les petits excès de vitesse ou encore de sanctionner lourdement l'usage de l'alcool et de stupéfiants au volant et les chauffards. Pour toutes ces raisons,

des ministères et des administrations qui, tous les soirs, avec des véhicules de fonction équipés de sirènes et de gyrophares, rentrent chez eux en toute illégalité, car non accompagnés d'un officier de police. La parole

le dossier de la sécurité routière est un sujet grave. J'en profite d'ailleurs pour me réjouir de la baisse de la mortalité sur nos routes depuis la fin de 2017,

Je souhaite dire ici qu'on ne répond pas à une mesure contre-productive par une autre mesure qui pourrait également l'être. Les médecins

c'est-à-dire appliquer les conclusions de notre rapport. J'ai donc quelque espoir qu'une parole tenue ainsi publiquement, après des mouvements aussi violents que ceux que notre pays a vécus, puisse enfin être tenue.

emmener la collectivité humaine qui nous est confiée vers un destin partagé en suscitant l'adhésion, bien évidemment de manière responsable. On peut aussi,

pays est confronté, que ceux qui sont dans la majorité méritent d'être soutenus, entendus, dans un esprit de responsabilité, sans céder nullement à la tentation populiste, à la démagogie ou à la seule défense d'un mouvement politique. Cela étant,

Selon l'exposé des motifs, cette mesure risquerait d'entraîner une augmentation des excès de vitesse. Curieux argument ... On peut aussi respecter la réglementation et ne pas commettre d'infraction ! Rappelons fortement que la route reste la première cause de mort violente en France

Quant à la vitesse, elle reste, qu'on le veuille ou non, la première cause d'accident mortel en France, suivie immédiatement- il est vrai -de l'alcool et des stupéfiants.

l'usage des stupéfiants et de l'alcool, en particulier. Il prévoyait également un certain nombre de dispositifs nouveaux en matière de prévention et de sensibilisation.

texte. Je pense en particulier au fait que la réduction du délai de récupération des points concernerait également les excès de vitesse commis en centre-ville ou sur les autoroutes, ainsi que d'autres infractions à la réglementation routière. Je ne crois pas que la déresponsabilisation des conducteurs soit l'objectif visé par cette proposition de loi. Notre objectif commun est bien de trouver un juste équilibre entre la lutte concrète contre l'insécurité routière et l'adoption de mesures qui ne soient pas ressenties comme injustes par nos concitoyens. Une réflexion sur la valorisation des comportements responsables sur la route est menée par le Conseil national de la sécurité routière. Ses conclusions devraient être présentées en ce début d'année. Attendons-les.

de la situation, cette proposition de loi est-elle la solution ? En effet, depuis le 1juillet, la vitesse maximale sur les routes à double sens, sans séparateur central, a été abaissée de 90 à 80 kilomètres Le code de la route prévoit que toute personne ayant perdu des points sur son permis de conduire les récupère automatiquement au bout de deux ans si elle n'a commis, dans ce délai, aucune nouvelle infraction au code de la route.

mois. Mes chers collègues, la sécurité routière ne se marchande pas. Il est question de vie humaine et de déplacements sécurisés. sécurisés. Parler sécurité routière aujourd'hui, c'est parler de vitesse, mais c'est aussi parler des infrastructures, car, ne nous y trompons pas, la sécurité tient beaucoup à l'état de ces infrastructures. L'entretien de la voirie coûte cher et incombe aux collectivités, qui n'ont pas de moyens suffisants. Classée première en 2011 pour l'état de ses routes, selon les critères du Forum économique mondial, la France n'est aujourd'hui plus que septième. C'est bien l'histoire d'une dégradation à la suite d'un manque d'investissement dans les infrastructures. La baisse des dotations de l'État aux collectivités, qui entretiennent les 370 000 kilomètres de routes départementales, comme la baisse des crédits pour les presque 12 000 kilomètres de routes nationales et d'autoroutes non concédées, se fait sentir sur les chaussées. Alors, à quelle suite Un nouvel ? Un #BalanceTonDépartement ou un #BalanceTaRouteDépartementale pour stigmatiser nos départements, qui n'ont plus les moyens d'assurer pleinement leurs compétences en la matière, comme vous avez pu le faire avec nos maires lorsque ces derniers ont dû augmenter les impôts locaux Les collectivités consacrent une part importante de leurs dépenses à la voirie. Elles représentent 9 % de celles des communes et plus de 8 % de celles des départements. la tendance générale est encore une fois à la baisse dans ce domaine. Il s'agit d'ailleurs d'une baisse considérable, puisque les dépenses de voirie des collectivités ont fléchi de 19 % entre 2013 et 2015. Cette orientation est confirmée par les premiers résultats publiés par l'Observatoire national de la route en novembre dernier. D'après l'analyse que je viens d'évoquer, laquelle a porté sur un échantillon de 57 départements, les chiffres montrent une baisse continue des dépenses de fonctionnement depuis 2013, qui touche tous les postes : les fournitures, notamment le sel pour la viabilité hivernale, la part de travaux confiée aux entreprises ou les frais généraux.

non prioritaires du réseau, ce qui pose des problèmes, non pas forcément en termes de bouchons, mais en termes de sécurité et de pérennité de voies qui n'ont pas été conçues initialement à cette L'état du réseau routier français se dégrade, et vous n'êtes pas sans savoir que la question du risque en matière de sécurité routière peut se poser. En cas d'accident, le défaut d'entretien peut entraîner la responsabilité de l'État. Investir sur nos routes est un vrai signal envoyé à nos concitoyens, le signal d'un État fort, soucieux de la sécurité des usagers de la route. Les Français n'ont pas besoin de panneaux limitant leur vitesse de plus ou moins 10 kilomètres par heure ; ils ont besoin de routes viables, sans nid-de-poule, salées en période de neige ; ils ont besoin de signalisation indiquant les zones réellement dangereuses. Ils n'ont surtout pas besoin de décisions prises de façon aléatoire, sans concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'heure où bon nombre de nos concitoyens occupent les routes et les ronds-points pour dénoncer un ras-le-bol général,

Cette mesure, entrée en vigueur le 1juillet dernier, a suscité la colère de nos élus et de nos concitoyens dans beaucoup de territoires. C'est un fait que les excès de vitesse les plus faibles sont les plus nombreux, et cela ne concerne pas uniquement la vitesse sur les routes secondaires. Aussi, lorsqu'ils sont flashés pour deux ou trois kilomètres par heure en trop, sommés de régler une amende et de perdre un point sur leur permis, beaucoup de nos concitoyens le vivent comme une injustice. Estimant que cette réduction de vitesse contribuera à faire « exploser » les amendes pour excès de vitesse inférieurs à 10 kilomètres par heure, les auteurs de la présente proposition de loi justifient dès lors de réduire le délai de récupération de points pour les petits excès de vitesse, en le faisant passer de six mois actuellement à trois mois, en l'absence de nouvelle infraction durant ce laps de temps. En outre, ceux-ci s'interrogent sur l'intérêt pédagogique du permis à points pour motiver ces aménagements. Je propose plutôt de nous interroger sur la portée de ce texte et sur sa réelle motivation. Sacrifier la sécurité routière au pouvoir d'achat n'est pas une bonne solution. Or modifier la procédure de récupération de points du permis de conduire va clairement à l'encontre de la politique de sécurité routière menée ces dernières années.

passer le délai de récupération de points à trois mois pourrait aisément inciter les conducteurs à relâcher leur vigilance et à ne plus se soucier de commettre un excès de vitesse, puisque le désagrément ne serait finalement que très bref. souvenez-vous que, avant 2011, il fallait attendre un an avant de récupérer le point perdu. Le passage de ce délai à six mois a été adopté contre l'avis du gouvernement et du ministre de l'intérieur de l'époque, Brice Hortefeux. Assouplir de nouveau ces règles à l'excès conforterait effectivement les mauvaises habitudes de conduite, même si elles ne concernent qu'une minorité de conducteurs. de loi stigmatisent en outre l'intérêt des stages de récupération de points, assimilés à une politique de sécurité routière répressive, et affirment que les points perdus ne sont jamais récupérés, sauf à effectuer- et donc à payer -un tel stage. Cela est faux. Certes, ces stages ont un coût financier et présentiel- c'est indéniable -, mais leur utilité en termes de prévention et de rétribution ne saurait être niée : quatre points en deux jours, tout de même ! Sans compter que cette récupération est automatique. Par ailleurs, le stage ne constitue pas la seule possibilité pour récupérer ses points. Il suffit d'attendre tout simplement la fin du délai de récupération sans commettre de nouvelle infraction, ce qui encourage les bons comportements sur les routes. Plus qu'un réel souci pour le pouvoir d'achat des Français, ce qui semble avoir motivé les auteurs de ce texte reste la dénonciation de la réduction de la vitesse à 80 kilomètres

que cette mesure avait renforcé le sentiment de déclassement de nos concitoyens qui n'ont pas d'autre choix que d'emprunter ces routes secondaires. Ce désaccord s'est traduit par la création au mois de janvier 2018 d'un groupe de travail sénatorial sur la sécurité routière, sur l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des lois. Plutôt que d'appliquer la réduction de vitesse de manière uniforme, ce groupe de travail a proposé que cette décision soit décentralisée au niveau des départements, afin de l'adapter aux situations locales et aux réalités des territoires. Cette conclusion convient à la plupart des maires et des élus. Je me félicite bien sûr que, à la suite du mouvement des « gilets jaunes », le Président de la République lui-même ait fait des annonces qui vont dans le même sens. En concertation avec les maires et les collectivités locales, l'application de cette mesure de réduction de la vitesse pourrait ne pas être généralisée, mais étudiée au cas par cas. Cependant, comme l'a dit mon collègue Michel Raison, il est vraiment dommage que les conclusions du groupe de travail sénatorial n'aient pas été entendues plus tôt par le Gouvernement. Cela aurait peut-être permis de ne pas cristalliser l'exaspération de nos concitoyens, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Cela démontre, s'il en était encore besoin, l'importance du travail sénatorial et la capacité du Sénat à trouver des solutions de compromis et de bon sens, qui respectent la diversité de nos territoires. Bien sûr, nous veillerons à ce que les annonces présidentielles soient suivies d'effets. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le secrétaire d'État. Cette proposition de loi me paraît donc désormais sans objet et, surtout, contre-productive en matière de sécurité routière, puisqu'elle va à l'encontre du principal intérêt pédagogique du permis à points, qui est d'inciter, de façon égalitaire, les conducteurs ne respectant pas les règles à modifier leur comportement sur la route pour ne pas perdre leur droit à conduire.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour débattre d'une proposition de loi particulièrement courte et simple : un article unique, une phrase, un mot changé dans le code de la route. Pourtant, ce texte apporte une avancée à la problématique du retrait de points pour infractions légères compte tenu, en outre, de la confusion sur certaines voies entre limitation de la vitesse à 80 kilomètres Un certain nombre d'amendements ont été déposés. On peut discuter de la pertinence ou non de chaque mesure, mais je note une chose en commun : l'ensemble de ces amendements visent à faciliter la vie des Français ou, du moins, à réduire les contraintes excessives de certaines réglementations. c'est bien là l'un des enjeux institutionnels que nous mettons aujourd'hui en exergue à travers ce texte : lorsque l'exécutif prend des mesures générales qui visent notre vie locale, elles complexifient et apparaissent souvent inopportunes ou insatisfaisantes. Face à cette réalité, le Sénat a une responsabilité particulière dans le cadre de nos institutions. Nous la connaissons bien : il s'agit de défendre nos territoires, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Le Gouvernement se donne deux ans pour évaluer la mesure. Nous gagnerions à engager notre propre évaluation. Il semble qu'il existe, et je conclurai par cette idée, une façon de concilier les différents objectifs avec celui- fondamental -de la réduction du nombre d'accidents sur nos routes, en modulant la limitation de vitesse à 80 ou 90 kilomètres par heure sur les routes secondaires en fonction de leurs caractéristiques.

et un ciblage de la limitation des vitesses maximales sur les routes accidentogènes. Dans l'attente d'une telle évolution, en souhaitant que la sécurité routière fasse toujours plus de pédagogie et de sensibilisation aux dangers de la route, je voterai en faveur de ce texte. va dans le sens d'une liberté accrue, ou au moins de contraintes réduites pour nos concitoyens de bonne volonté, sans remettre en cause l'objectif fondamental de la sécurité routière. Je l'espère vivement, il y aura moins de conducteurs privés de permis de conduire qui font la folie de prendre tout de même la route pour ne pas perdre leur emploi, ce qui est un véritable drame pour notre société.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat qui nous rassemble est l'occasion de tirer les enseignements d'un processus de décision qui illustre une méthode de gouvernement méritant sans doute d'être affinée. Sous couvert de lutter contre la mortalité routière, le Gouvernement a annoncé vouloir abaisser la vitesse à 80 kilomètres par heure sur toutes les routes, et ce sans étude d'impact ni concertation. Des voix se sont élevées ici et là, singulièrement au Sénat, pour demander des explications et proposer de laisser des possibilités d'adaptation aux acteurs locaux. Je pense en particulier à nos collègues Raison, Vullien et Fichet. Le Premier ministre n'a rien voulu entendre. Le décret a été signé et a dû s'appliquer sans délai. Tous ceux qui émettaient des réserves ont été vilipendés au nom de la mortalité routière et passibles de procès en irresponsabilité.

Alors que la réduction de la dépense publique est un objectif, on peut s'interroger sur l'évaluation qui a pu être faite du coût de cette mesure, tant pour les services publics que pour les entreprises et les salariés. salariés. La question de l'acceptabilité et de la compréhension par les usagers de la route qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler est taboue. Les experts savent et le Gouvernement décide. J'ai envie de dire : « Circulez, il n'y a rien à voir ! » Je pense très sincèrement, monsieur le secrétaire d'État, que cette mesure a contribué à faire émerger le mouvement des « gilets jaunes », car elle est emblématique, dans la forme comme sur le fond, d'une pratique qui conjugue suffisance, suffisance, mépris des réalités, jacobinisme et autoritarisme. On le sait, la politique n'est pas une science exacte et ce qui compte est souvent davantage la perception de la mesure que sa justification. On ne gouverne pas un pays sans explications et avec les seuls experts contre l'opinion. L'humilité, permettez-moi de vous le dire, loin d'être un signe de faiblesse, peut quelquefois être un signe d'intelligence. Aujourd'hui, un texte nous est soumis pour apporter une réponse à une situation que beaucoup récusent et vivent comme une brimade. Merci aux auteurs de cette proposition de loi d'avoir posé le débat publiquement ! Je ferai trois remarques plutôt que de chercher à agir sur les conséquences d'une mauvaise décision, je pense préférable d'agir sur la décision elle-même, et donc de revenir tout simplement sur le décret. le décret. Ensuite, nous avons l'illustration de la difficile articulation entre le décret et la loi. C'est un décret qui est à l'origine de la situation. On ne corrige pas un décret par une loi. Le décret procède de la loi et non l'inverse. Cela ne peut que nous conforter dans notre regret de voir le Gouvernement, dans cette affaire comme dans bien d'autres, refuser le débat au Parlement et passer outre ses avis. Nous écouter lui aurait évité ce faux pas. c'est avec étonnement que nous avons entendu le Président de la République déclarer la semaine dernière qu'il n'était pas hostile à une évolution de la réglementation. Feignant de découvrir le sujet, c'est tout juste s'il n'a pas fait le reproche aux parlementaires de ne pas l'avoir alerté sur ce point. Cela ne manque pas de piquant si l'on se réfère aux propos tenus ici même par Michel Raison lors d'une question d'actualité au Gouvernement et

pour les retraits de points au permis de conduire. Il s'agit de prévoir qu'aucun retrait de points ne peut être appliqué à une personne plus de trois ans après la commission d'une infraction. En l'état du droit, le retrait de points s'applique à compter du jour où la condamnation est devenue définitive et non à compter de la date à laquelle le courrier informant d'un retrait de points est reçu par le détenteur du permis. Par exemple, si une personne commet un excès de vitesse constaté par un radar automatique, le retrait de points s'applique à compter du moment où la personne a payé son amende. Il n'est donc pas nécessaire d'encadrer davantage les règles en matière de retrait de points, dont les principes sont déjà clairement énoncés par la loi. J'émets donc un avis défavorable

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

du Gouvernement, tout en rappelant, naturellement, l'importance de se comporter de manière responsable sur la route. La structure des vitesses maximales autorisées sur certains tronçons routiers a été terriblement

sur l'ensemble de nos routes, soit on revient sur la question du permis à points. Dans tous les cas, c'est un autre débat que celui qui est posé ici. La parole est à M.

d'instaurer un sursis pour le retrait de point dans le cas d'excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure commis sur les routes limitées à 80 kilomètres par heure. Cet amendement n'est pas sans intérêt, car il vise à valoriser les comportements les plus vertueux sur la route et à ne pas pénaliser démesurément les conducteurs les plus responsables.

Surtout, compte tenu de la complexité de la matière, il paraît préférable de conditionner toute évolution législative du permis à points à la réalisation d'une étude d'impact approfondie,

Le scrutin est ouvert.

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie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

madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la qualité de vie des personnes âgées et l'accompagnement de la perte d'autonomie sont deux priorités que s'est fixées le Gouvernement. Comme vous tous, nous sommes convaincus que mieux prendre en charge nos aînés est un devoir de solidarité. Plusieurs réformes sont déjà en cours pour avancer vers une société plus inclusive et protectrice pour les personnes âgées. Je pense en particulier à la transformation du système de santé autour du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques, aux nouvelles synergies entre médecine de ville, secteur médico-social et hôpital et à la suppression progressive du reste à charge pour les assurés dans les domaines de l'optique, du dentaire et de l'audiologie. Cette dernière réforme, majeure, répondra aux attentes des personnes âgées, qui auront plus facilement accès à un ensemble de prestations de soins identifiées et nécessaires : bien voir, bien entendre et soigner son hygiène bucco-dentaire. Concrètement, depuis le 1 janvier, la base de remboursement des aides auditives est passée de 200 à 300 euros, soit 200 euros de reste à charge en moins par oreille. Dès 2020, l'absence de reste à charge sera garantie en optique et sur une partie du panier dentaire : les couronnes et les bridges. L'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées passe aussi par une transformation en profondeur de la manière dont est reconnu et pris en charge le risque de perte d'autonomie lié au vieillissement. Comme vous le savez, le Gouvernement a lancé en octobre dernier une vaste concertation et un débat national autour du grand âge et de la perte d'autonomie. Cette mission, conduite par Dominique Libault, formulera des propositions d'ici au mois de mars, afin de couvrir l'ensemble des aspects de la prise en charge des personnes âgées. Un projet de loi sera ensuite déposé devant le Parlement. Sans remettre en cause ces différents travaux, qui s'inscrivent sur le temps long, la proposition de loi soumise à votre examen vise à répondre à un problème précis et concret : l'accès aux soins ophtalmologiques dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

Des mesures ont été prises pour étendre les champs de compétence des orthoptistes et des opticiens-lunetiers, mais, chacun en convient, elles n'ont pas résolu l'ensemble des problèmes. L'article unique de la proposition de loi visait initialement à lever une restriction, afin de permettre aux personnes âgées hébergées en EHPAD de bénéficier d'un test de réfraction et d'une adaptation de leur correction sans avoir à se déplacer chez un opticien. Néanmoins, si les préoccupations sont légitimes et partagées, il est compliqué de légiférer sur ce sujet sans s'assurer au préalable que les conditions de qualité et de sécurité des soins sont réunies. Or, chez le patient âgé, les pathologies oculaires, qui peuvent se traduire par une baisse de l'acuité visuelle, sont fréquentes et nombreuses. Seul un examen ophtalmologique complet permet de les détecter, un examen que l'opticien n'est pas en mesure de faire. Pour cette raison, le Gouvernement appuie la position adoptée par l'Assemblée nationale, qui privilégie la voie de l'expérimentation. Le texte prévoit ainsi d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser directement dans les EHPAD une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales. Cette expérimentation n'étend donc pas les compétences des opticiens-lunetiers ; elle leur permet seulement de délocaliser l'exercice de leur activité au plus près de personnes ne pouvant se déplacer. J'ai entendu les critiques qui se sont exprimées en commission sur le manque d'ambition de ce texte. Cette proposition de loi a été déposée par le groupe UDI, Agir et Indépendants. Le Gouvernement y apporte un soutien que je qualifierai de pragmatique, il ne s'agit nullement d'éluder le sujet plus large de l'accès aux soins. Je rejoins les propos que vous avez tenus la semaine dernière en commission : nous devrons ouvrir le chantier plus large de l'organisation de la filière visuelle. Pour répondre aux difficultés d'accès aux soins dans les territoires, il nous faut également nous appuyer davantage sur le numérique. C'est le sens de l'entrée dans le droit commun des pratiques médicales de la télémédecine en 2018. La téléconsultation est ainsi remboursée par l'assurance maladie depuis le 15 septembre dernier, à l'instar des consultations classiques. Nous héritons d'une démographie médicale en souffrance, et les décisions louables sur le mettront plusieurs années à porter leurs fruits. Aussi toutes les solutions doivent-elles être explorées. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé se construit dans le souci de structuration des soins de proximité et de constitution d'un collectif de soins. Des ponts et des outils de coopération doivent être créés entre hôpital, ville et secteur médico-social. Nous sommes convaincus que l'exercice coordonné a vocation à se développer,

la commission des affaires sociales a examiné le 16 janvier dernier, en application de la procédure de législation en commission, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale sur l'initiative du groupe UDI, Agir et Indépendants, relative à la santé visuelle des personnes âgées hébergées en établissement. L'adoption conforme de ce texte et sa promulgation prochaine ouvriront à l'opticien-lunetier la possibilité d'accomplir dans l'établissement un test de réfraction de l'acuité visuelle

Bien qu'elle ait adopté cette proposition de loi, qui apporte un assouplissement bienvenu à la pratique des soins optiques destinés aux personnes âgées, la commission des affaires sociales n'a pas manqué de faire part à Mme la secrétaire d'État des attentes immenses qui subsistent en matière d'accès aux soins visuels. Offrir Offrir la possibilité aux opticiens d'exercer leur art en établissement est, sur le papier, un indéniable progrès. Je crains néanmoins que l'effet de cette mesure ne se révèle dans les faits particulièrement limité. limité. En effet, la possibilité pour l'opticien d'adapter l'équipement optique d'une personne âgée restera conditionnée à la production par cette dernière d'une ordonnance délivrée par un ophtalmologiste moins de trois ans auparavant. Or nous savons tous que, du fait des difficultés d'accès de la population à des soins ophtalmologiques très contraints par la démographie médicale, cette condition de délai est rarement remplie au moment d'une entrée en EHPAD. En conséquence, le nouveau droit ouvert risque fort de ne pas trouver à s'appliquer. Indubitablement, le vrai problème, auquel cette proposition de loi ne répond pas, demeure celui de l'accès au prescripteur médical. Comme déléguée à l'accès aux soins auprès de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, je suis intimement convaincue que le principal défi aujourd'hui posé au législateur concerne la délégation d'actes médicaux. le principal défi qui se pose aux territoires supposera d'impliquer tous les professionnels de la santé visuelle. La pénurie croissante de l'offre de soins en ophtalmologie a provoqué la mobilisation

La loi de modernisation de notre système de santé, dont j'avais assuré le rapport au côté de notre président, Alain Milon, et de ma collègue Catherine Deroche, avait redéfini les termes de leur collaboration avec les ophtalmologistes, afin de leur permettre d'accomplir les actes médicaux de premier recours. Bien que porteuse d'indéniables progrès, cette loi doit être retravaillée et approfondie, afin que la filière visuelle s'approprie pleinement les possibilités nouvelles offertes, notamment, par la télémédecine. En l'état actuel de notre droit, et malgré l'adoption de la présente proposition de loi, je crains fort que l'équipement optique des personnes âgées accueillies en établissement ne continue à pâtir d'une offre de soins faiblement accessible et inégalement distribuée sur le territoire national. Un autre regret me vient des modifications apportées par l'Assemblée nationale en séance publique au texte initialement conçu par ma collègue députée Agnès Firmin Le Bodo.

Dans la mesure où ces conventions sont déjà incluses dans le contrôle de qualité externe auquel les EHPAD sont obligatoirement soumis depuis la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, je considère cette précaution comme superflue au lieu de protéger la personne, elle risque de la priver de l'opportunité offerte par ce texte. Plusieurs membres de la commission des affaires sociales, auxquels je me joins, se sont également émus de ce que l'adoption d'un texte aussi modeste révèle de l'importance de l'initiative parlementaire

Pour cela, elle prévoit d'ouvrir la possibilité, pour les opticiens, de se déplacer dans les EHPAD en vue de réaliser sur place des tests d'acuité visuelle, et de déceler la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Ce texte vise à répondre à deux problèmes sous-jacents qui touchent les personnes âgées : les pertes de mobilité et la forte prévalence des troubles de la vue au sein de cette population. Pour faire face à la pénurie d'ophtalmologistes, les opticiens sont habilités à pratiquer des examens pour mesurer la vision et délivrer un équipement adapté, mais seulement dans leur magasin

Cela est encore plus vrai en EHPAD où les pensionnaires, souvent très dépendants, ne peuvent se rendre chez l'opticien, le transport n'étant pas pris en charge. Pourtant, nous savons que le dépistage et la correction des troubles visuels constituent un point important dans la préservation de l'autonomie et de la qualité de vie.

Les opticiens proposent d'améliorer l'accès à la santé visuelle des résidents en EHPAD en pratiquant des examens pour dépister les troubles de la réfraction et engager des actions de prévention et d'accompagnement de la santé visuelle Nous mesurons l'importance d'adopter cette proposition de loi conforme. Cependant, il serait souhaitable d'y associer un dispositif d'information destiné au médecin traitant, visant à l'informer des résultats de l'examen mis en oeuvre par l'opticien, en particulier lorsque des troubles de la réfraction ou des troubles associés ont été détectés, et de la nécessité d'une consultation ophtalmologique. Il serait également judicieux de permettre aux orthoptistes de pratiquer leurs examens en EHPAD sous l'autorité d'un ophtalmologiste. Cette proposition de loi prévoit de lever le frein d'accès aux soins visuels de nos aînés qui résident en EHPAD concernant les troubles de réfraction. Notre groupe soutient cette avancée importante pour nos aînés en EHPAD, malgré la restriction de son application aux seules ordonnances de moins de trois ans de l'ophtalmologue. Plus généralement, dans le cadre des travaux sur la perte d'autonomie, l'amélioration du parcours de soins et de la qualité

La France se caractérise par un taux élevé en EHPAD : 40 % des personnes âgées en perte d'autonomie. Des mesures de maintien à domicile doivent être améliorées en faveur des aidants, en revalorisant les salaires des intervenants, en augmentant les SSIAD, en mettant en place de l'accueil de jour, mais l'hébergement en EHPAD restera incontournable : grande dépendance, personnes seules, troubles cognitifs. Le personnel soignant- aides-soignantes, infirmières -devra être augmenté, et donc la dotation soins aux EHPAD majorée pour avancer vers un encadrement plus important, préalable à une prise en charge décente de nos aînés. décente de nos aînés. Si la sécurité sociale est à l'équilibre et la CADES remboursée en 2024, il y aura, à ce moment, une possibilité de financement qui pourrait être affecté aux personnes âgées. Toutefois, madame la secrétaire d'État, dès 2020, il faudra augmenter les dotations soins aux EHPAD de façon sensible. Madame la secrétaire d'État, nous attendons votre annonce prochaine du projet de loi sur l'autonomie, qui devra, nous l'espérons, replacer la prise en charge des personnes âgées, notamment dépendantes, au centre de la société, avec une solidarité digne de nos aînés. En attendant, notre groupe votera bien sûr la proposition de loi.

la France compte aujourd'hui 1,5 million de personnes de quatre-vingt-cinq ans et plus. En 2016, près de 7 500 EHPAD accueillaient 608 000 personnes. Ces chiffres donnent la mesure des enjeux concernant le vieillissement de la population. Le dispositif actuel ne permet pas aux personnes accueillies en EHPAD de disposer de lunettes adaptées à leur correction. L'obtention d'un rendez-vous avec un ophtalmologue est actuellement de 80 jours en moyenne. Cela s'avère encore plus compliqué pour les personnes âgées en établissement. Cette situation risque encore de s'aggraver dans les années à venir. En 2030, la densité moyenne d'ophtalmologues libéraux devrait s'élever à six médecins pour 100 000 habitants, soit une diminution de 20 % par rapport à 2016. Ces difficultés d'accès à une consultation ophtalmologique sont donc appelées à perdurer. De surcroît, les personnes âgées portent trop souvent des lunettes inadaptées : des chercheurs de l'INSERM ont publié récemment une étude qui montre que près de 40 % d'entre elles souffrent d'un trouble visuel mal corrigé. L'altération de la vue a une incidence directe sur l'autonomie et la sécurité des personnes âgées, car elle se répercute sur le risque de chutes, l'isolement et la perte d'autonomie. Enfin, les difficultés de mobilité des personnes âgées compliquent l'accès à des consultations en dehors de l'EHPAD. À la suite de ces différents constats, cette proposition de loi permettra d'offrir la possibilité aux opticiens-lunetiers de pratiquer des tests de réfraction et des adaptations de verres correcteurs ou de lentilles de contact au sein des EHPAD. La correction de la vue doit d'abord être prescrite par un ophtalmologue, la prescription peut ensuite être adaptée par un opticien-lunetier. Cette adaptation est effectuée dans le cadre d'une opération dite « de réfraction au cours de laquelle le professionnel mesure le défaut optique et détermine la qualité de l'équipement à fournir. Depuis 2007, les opticiens sont autorisés à réaliser des tests d'acuité visuelle dits de « réfraction » afin d'adapter les ordonnances délivrées par les ophtalmologues. Toutefois, cette proposition de loi ne concerne que les modalités de renouvellement de l'équipement optique des personnes hébergées en établissement. De plus, la portée de ce texte a malheureusement été restreinte à la suite de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de réécriture de son unique article. Cette réécriture a limité de manière excessive la possibilité d'intervention de l'opticien-lunetier en EHPAD en soumettant cette possibilité à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier ne pourra y recourir que dans un cadre expérimental et pour une durée de trois ans. Cette réécriture limite la désignation de quatre régions au plus dans lesquelles l'expérimentation pourra être menée. Ainsi, une fois que les quatre seules régions auront été déterminées, la mise en oeuvre de cette proposition de loi sera revêtue d'un caractère expérimental, et ce texte réservera au directeur général de l'ARS concernée le pouvoir de ne pas l'autorisation d'intervention de l'opticien-lunetier en EHPAD. Ces restrictions excessives risquent d'entraver sérieusement la mise en oeuvre de ce texte. C'est tout à fait regrettable ! Il est dommage également que le champ de cette proposition de loi n'ait pas été élargi, alors qu'il s'agissait d'une opportunité pour étendre aux personnes âgées en EHPAD l'accès aux soins auditifs. Enfin, ce texte aurait pu s'inscrire dans une vision d'ensemble de réorganisation de la filière visuelle. Améliorer la prise en charge des personnes âgées est un devoir de solidarité. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera en faveur de cette proposition de loi, en regrettant toutefois son manque d'ambition et les restrictions apportées par l'Assemblée nationale.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, déposée par la députée Agnès Firmin Firmin Le Bodo. Je me félicite que le groupe Union Centriste au Sénat ait choisi de reprendre le texte, qui fait l'objet d'un consensus transpartisan, en améliorant la vie quotidienne de nos aînés. de loi permet de mieux prendre en compte la dépendance des personnes âgées en EHPAD et de tendre vers l'objectif d'un suivi médical accessible à tous les publics. Elle répond à une problématique réelle. Nombreux sont les résidents en EHPAD qui pâtissent d'un équipement optique inadapté à leurs besoins. Une récente étude de l'lNSERM Alienor indique que 40 % des sujets âgés de plus de soixante-dix-huit ans n'ont pas de lunettes adaptées à leur vue. De plus, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie est aujourd'hui de cinquante-deux jours. À cette attente importante s'ajoute la difficulté de se déplacer des personnes en EHPAD, chaque rendez-vous nécessitant un accompagnement qui n'est pas aisé à mettre en oeuvre. Or la santé visuelle des personnes âgées ne doit pas être perçue comme secondaire. D'une part, comme pour chacun d'entre nous, elle est essentielle pour mener à bien toutes les activités du quotidien d'autre part, elle permet de réduire des risques graves auxquels nous sommes particulièrement exposés à un âge avancé, tels que les chutes, qui ont souvent des conséquences fatales. Enfin, autre point non négligeable, la vue est un vecteur de sociabilité. Le rapport MONALISA- Mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés -montre que la France est le troisième pays d'Europe le plus touché par le problème de l'isolement

L'impact de la solitude chez les personnes âgées peut être dévastateur, avec des dommages qui affectent tout le corps. L'isolement social est un aspect à prendre en compte dans l'évaluation clinique d'un patient âgé. En fait, la solitude représente un facteur de risque important pour l'altération de la fonction cognitive des personnes âgées. L'objectif du présent texte, que le groupe La République En marche partage, est donc d'accompagner au mieux la perte d'autonomie des personnes en EHPAD, pour éviter d'accroître davantage leur dépendance. Concrètement, cette proposition de loi doit permettre aux opticiens-lunetiers de venir à la rencontre des personnes qui en ont besoin. Rappelons qu'elle n'étend pas les compétences de ces derniers, qui ont déjà la possibilité de réaliser des tests d'acuité d'acuité visuelle dits de « réfraction » dans leurs boutiques depuis 2017 ; mais elle délocalise leur exercice au plus près des personnes ne pouvant pas se déplacer. La proposition de loi maintient également l'obligation d'une consultation médicale en ophtalmologie datant de moins de trois ans et s'inscrit, en outre, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et de la mise en place du reste à charge zéro. zéro. Une telle expérimentation sera sans aucun doute bénéfique pour de nombreux résidents en EHPAD, dans un souci de prise en compte de leur situation de dépendance et dans le sens d'une plus grande fluidité du parcours de soins visuels. Elle est d'ailleurs particulièrement sensée en milieu rural, où l'accompagnement est difficile à mettre en place. Enfin, elle participe à l'objectif du Gouvernement depuis le début de ce quinquennat, avec le programme « 100 % santé », à savoir favoriser l'accès aux soins, notamment pour les assurés sociaux les plus démunis,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à titre liminaire, je regrette le recours, une fois de plus, à la procédure en commission, qui prive les textes de débats publics. Alors même que nos concitoyennes et concitoyens contestent nos institutions et demandent davantage de démocratie, de transparence sur les prises de décisions politiques, la majorité sénatoriale choisit cette procédure qui laisse les débats se dérouler en commission au détriment de la séance publique. À cela s'ajoute la pression du Gouvernement pour que nous adoptions conforme ce texte afin de garantir son application rapide, au détriment des prérogatives des parlementaires que nous sommes. À l'heure où les « gilets jaunes » réclament davantage de démocratie avec la création du référendum d'initiative citoyenne et critiquent la démocratie représentative, le recours à la législation en commission et l'exigence de ne pas amender ce texte sont un mauvais signal envoyé, d'autant que nous en avons des choses à dire sur l'accès aux soins des personnes âgées dépendantes ! Or la proposition de loi de notre collègue députée Agnès Firmin Le Bodo, examinée aujourd'hui, apporte une réponse très limitée, en autorisant les opticiens à se rendre dans les EHPAD pour contrôler l'acuité visuelle des personnes. L'Assemblée nationale a modifié ce texte en une simple expérimentation des opticiens-lunetiers à délocaliser leur exercice au profit des personnes ne pouvant se déplacer. Le secteur mercantile de l'optique va pouvoir se satisfaire de ce nouveau texte, qui s'ajoute aux libéralisations de la profession déjà en cours et au déficit chronique d'ophtalmologues. Ainsi, plutôt que de chercher des solutions aux carences de professionnels de santé, ce texte propose une sorte de rustine en autorisant les opticiens-lunetiers à les remplacer partiellement. Il s'inscrit dans le droit fil de la loi Croissance et activité de 2014, dite « loi Macron », qui tendait à supprimer l'obligation d'ordonnance pour les verres correcteurs, et du décret du 12 octobre 2016, qui autorise les opticiens à à adapter les prescriptions médicales des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices lors d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction. Autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser des examens de réfraction dans les EHPAD est une solution simpliste qui ne répond pas aux racines du problème, à savoir le nombre insuffisant d'ophtalmologistes sur notre territoire et les difficultés d'accès aux soins. Nous regrettons d'ailleurs que ce texte se limite aux difficultés d'accès aux soins d'optique alors que les les inégalités territoriales et les déserts médicaux concernent l'ensemble des généralistes et des spécialistes. La santé visuelle des personnes dépendantes est un sujet très important, et, comme tous nos collègues, nous ne pouvons accepter que 40 % des personnes âgées de plus de portent des lunettes non adaptées à leur vue. Nous savons que, pour une proportion importante d'entre elles, les difficultés financières expliquent les renoncements à modifier leurs lunettes. En réalité, loin de résoudre les problèmes, vous allez prendre le risque d'en créer de nouveaux, en faisant entrer les opticiens dans les EHPAD. Ainsi, quelles garanties pouvez-vous nous apporter afin d'entourer, d'accompagner des personnes personnes âgées dépendantes et naturellement fragiles face à des commerciaux intéressés à vendre leurs lunettes ? Nous ne contestons pas l'importance du métier d'opticien-lunetier, qui se vérifiera encore davantage avec le vieillissement de la population et l'utilisation des écrans. Cependant, les ophtalmologues doivent demeurer la porte d'entrée pour les soins d'optiques. Alors que le nombre d'ophtalmologues a diminué de 5,7 % entre 2007 et 2017 selon la DREES, il faut inverser la tendance. Nous proposons donc de supprimer le des ophtalmologues comme le Gouvernement l'a fait pour les médecins. C'est d'ailleurs le souhait du président du Syndicat national des ophtalmologistes de France, Thierry Bour : « Débloquer le quota des postes d'internes serait une mesure très efficace, car 100 % des postes produisent un ophtalmologiste diplômé cinq ans plus tard. » Il est donc indispensable pour mon groupe de revaloriser la profession d'ophtalmologues et de favoriser les installations dans des centres de santé publics accessibles dans chaque canton, afin de lutter contre les inégalités territoriales. loi de financement de la sécurité sociale, que les frais d'optique prescrits soient pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. C'est d'une tout autre logique que votre « 100 % santé », qui, comme nous l'avions dénoncé sans trouver d'écho auprès de Mme la ministre de la santé, Agnès Buzyn, se répercute auprès des assurés par une augmentation des mutuelles. Nous regrettons enfin que le texte reste muet sur le fait que les personnes en perte d'autonomie ne puissent consulter facilement un professionnel de santé par par manque de personnels dans les EHPAD. En attendant de débattre avec la ministre de la santé de son projet de réorganisation de notre système de santé, qui répond peut-être positivement à certaines de nos propositions que j'ai brièvement exposées- on ne sait jamais, je peux formuler quelques voeux

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, est d'effet limité. Toutefois, elle est porteuse d'améliorations concrètes pour certains de nos concitoyens âgés. Dans le prolongement du décret d'octobre 2016, ce texte relève d'un objectif simple : apporter une réponse aux difficultés d'accès aux soins visuels de nos aînés, en prévoyant d'autoriser les opticiens

loi permettrait donc de limiter- un peu -les effets du nombre insuffisant d'ophtalmologistes et d'améliorer la santé visuelle des personnes dépendantes. L'accès aux soins visuels représente un défi démographique en France.

Cette proportion élevée s'explique tant par des difficultés financières que par une forme de fatalisme des personnes en perte d'autonomie à l'égard des troubles de la vision, lesquels s'aggravent naturellement avec l'âge.

Or, comme les troubles de l'audition, une vue déficiente produit des effets néfastes sur la santé d'une personne âgée. Elle se répercute sur sa qualité de vie et sur son autonomie, induisant une marche hésitante, des risques de chute, une La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui remédie en partie à cette situation. La réalisation d'examens visuels dans les EHPAD épargnerait aux aidants ou au personnel soignant de devoir déplacer les personnes en perte d'autonomie vers des lieux éloignés en vue d'une consultation ou de soins. Pour les opticiens, ce nouveau droit complète l'autorisation octroyée par le décret du 12 octobre 2016, qui leur permet d'adapter les prescriptions médicales des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction. Mais, dans le cadre réglementaire actuel, ces examens doivent être réalisés dans un espace adapté, afin de garantir de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, dans un magasin d'optique-lunetterie. de loi est restreinte : elle ne s'inscrit pas dans une vision globale de réorganisation de la filière visuelle ; elle n'apporte pas non plus de solutions aux problèmes structurels d'accès aux soins visuels sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, les membres du groupe socialiste et républicain partagent le diagnostic

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis pour voter la proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées : un intitulé ambitieux pour un texte qui, à mon grand regret, suscite quelque frustration, y compris dans les rangs du groupe RDSE. Ce manque d'enthousiasme a bien sûr trait au contenu de la proposition de loi, et non à sa thématique : sur le fond, nous sommes nombreux, au sein de cette assemblée, à être très préoccupés par les inégalités d'accès aux soins, qu'elles soient sociales ou territoriales.

Les problèmes systémiques de la filière sont connus et appellent des réformes profondes. Le plan de transformation du système de santé qui sera présenté dans les prochains mois a au moins partiellement vocation, je l'espère, à répondre à la pénurie de praticiens.

personnes doivent être accompagnées par des membres du personnel soignant -or, en EHPAD, ces derniers ne sont pas toujours disponibles -ou faire appel à la solidarité familiale, ce qui n'est pas toujours possible non plus, compte tenu des situations d'éloignement. Ces déplacements sont donc un frein réel à l'accès aux soins.

de soins et de respect des normes. Nous parlons ici de structures dans lesquelles les résidants sont accompagnés par du personnel soignant à même d'organiser ce service dans de bonnes conditions. Pour ma part, j'irai encore plus loin, en proposant de réfléchir à une généralisation de la mesure à toutes les personnes âgées, quel que soit leur lieu de résidence. Une telle même si nous n'étions pas en situation de pénurie de praticiens, pourquoi imposer à nos aînés des déplacements inutiles ? En leur permettant de rester sur leurs lieux d'habitation ou de résidence, comme les EHPAD, on limite les contraintes qui les éloignent des soins et l'on favorise, tout simplement, des conditions de consultation plus sereines.

? Les demandes de visites augmentant avec le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie, certains opticiens se rendent déjà à domicile pour présenter leurs équipements. Nous savons bien que, à cette occasion, des tests sont effectués. proposition de loi permettra de sécuriser juridiquement cet examen réalisé en EHPAD. Ne pourrait-on pas aller plus loin, au moins étudier les conditions dans lesquelles les opticiens pourraient également rendre visite aux personnes âgées qui demeurent à leur domicile ? Rappelons qu'il ne s'agit pas là d'une extension de compétences, mais d'une simple délocalisation de l'activité. La désertification des territoires et le vieillissement de la population nous obligent à revoir totalement les pratiques des professionnels, à les réinventer, à nous libérer des carcans d'un autre temps pour innover. occasion pour évoquer de nouveau la question des transports hospitaliers. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, nous sommes nombreux à avoir alerté le Gouvernement sur les difficultés financières rencontrées à la fois par les établissements et par les petites entreprises de transport.

Ainsi, c'est souvent dans une situation de santé dégradée que le placement est décidé. Au regard de ce défi toujours plus grand pour les EHPAD, il convient d'assouplir notre droit. Les améliorations que nous pouvons apporter permettront d'améliorer la qualité de vie

l'on oeuvre dans ce sens, la personne est gagnante et la qualité de vie dans l'EHPAD s'en ressent. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail de notre collègue députée Mme Firmin Le Bodo, auteur de cette proposition de loi.

d'une autorisation de l'ARS complexifie davantage encore la démarche. Si nous soutenons habituellement le recours aux expérimentations, nous ne pouvons, en l'espèce, que nous en alarmer.

Or le Gouvernement n'a de cesse de nous rappeler qu'il travaille aujourd'hui à un grand texte sur la dépendance : la rédaction de ce projet de loi, la remise de l'avis du Conseil d'État, puis la navette parlementaire auraient constitué autant de moments opportuns pour adapter le dispositif que nous aurions pu adopter dès aujourd'hui. de la proposition de loi initiale prive donc de nombreuses personnes d'une amélioration importante de leur qualité de vie. Je regrette que l'exécutif n'ait pas opté pour une démarche d'amélioration continue, rendue possible par l'agenda du Gouvernement, plutôt que pour le recours à une expérimentation nécessairement inégalitaire entre les territoires. Pour tous les sujets relevant de la dépendance, il pourrait être opportun d'envisager l'adoption des mesures figurant à l'agenda du Parlement, afin que les retours d'expérience viennent abonder la rédaction du futur projet de loi pour améliorer,, sa portée et sa justesse. Parler de la santé de nos anciens, de leur qualité de vie en EHPAD, de l'accompagnement que nous pouvons leur offrir, c'est parler de notre propre avenir ; c'est parler en fait de notre société et de la solidarité intergénérationnelle que nous souhaitons.